Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 7 juin, après la séance de questions d'actualité au Gouvernement, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs. Acte est donné de cette demande. La commission des affaires économiques se réunira le mardi 6 juin, à neuf heures trente, pour l'examen du texte et du rapport. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé au mercredi 7 juin, à onze heures, et le délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale, au mardi 6 juin, à quinze heures. Y a-t-il des observations ?

à la détection des mouvements de véhicules ou d'événements prédéterminés, la version initiale du projet de loi est plus précise, puisqu'elle vise « l'identification des infractions précitées ». Il doit être entendu que les critères de recherche qui seront définis par décret en Conseil d'État et qui seront exploités par les agents destinés exclusivement à détecter des mouvements susceptibles de révéler les infractions visées au premier alinéa de l'article 11 du présent projet de loi.

professionnel, mais ils ont été désignés en qualité de gardes-frontières à la Commission européenne au sens du code frontières Schengen. Ils exercent par ailleurs sur le territoire des contrôles de titres d'entrée et de séjour en zone frontalière.

que vous proposez semble impliquer que les agents de douane judiciaire seront désignés et nommés par des magistrats, ce qui n'est pas le cas des officiers de douane judiciaire.

monsieur le ministre.

vise à responsabiliser les plateformes de partage de contenus en ligne quant à leur participation de fait à l'essor du commerce parallèle illicite de tabac, en limitant le

et à augmenter les peines encourues par les trafiquants de tabac, ce qui permettra de maintenir la hiérarchie entre les infractions simples et en bande organisée, tout en tenant compte de la spécificité criminologique des trafics

Monsieur le ministre,